La séance est reprise. Mes chers collègues, en raison de la tenue de la Conférence nationale des territoires, et en accord avec les commissions concernées et le Gouvernement, le début de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2017, initialement prévu jeudi 14 décembre, à dix heures trente, devrait être fixé le même jour, à Le délai limite de dépôt des amendements sur ce texte resterait fixé à dix heures trente. En conséquence, la discussion de la proposition de résolution visant à pérenniser et adapter la procédure de législation en commission, présentée par M. Gérard Larcher, président du Sénat, serait inscrite à l'ordre du jour du matin, à dix heures trente. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable- vingt-neuf voix pour, zéro voix contre et trois bulletins blancs -à la reconduction de M. Jean Bassères aux fonctions de directeur général de Pôle emploi. emploi. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2018. Nous poursuivons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Cohésion des territoires » (et articles 52, 52 bis, 52 ter, 52 quater, 52 quinquies et 52 sexies).

nous examinons cet après-midi les crédits d'une nouvelle mission, « Cohésion des territoires », qui regroupe les crédits de deux précédentes missions, « Égalité des territoires et logement » et « Politique des territoires

d'aborder quelques points saillants, et il y en a cette année ! La mission constitue tout d'abord l'un des principaux postes d'économie du budget général, puisqu'elle connaît la plus forte baisse de crédits de paiement en un an, soit 1,7 milliard d'euros. Cette tendance se poursuivra également sur le plan triennal 2018-2020, avec une diminution de 8,3 % en valeur, tandis que les crédits du budget général augmenteront parallèlement de 3 %. Cette baisse en 2018 de la dépense publique de l'État est principalement supportée par le programme 109, qui finance les aides personnelles au logement, les APL, et voit son enveloppe se réduire de 1,9 milliard d'euros.

Surtout, nous aurons l'occasion d'y revenir longuement lors de l'examen de cet article, derrière une prétendue mesure en faveur du pouvoir d'achat des locataires, qui sera dans les faits très minime, malgré des effets d'aubaine pour certains, et une réforme de structure des organismes de logement social, vous proposez en réalité une mesure de rendement budgétaire permettant de réduire la dépense publique.

La baisse des aides personnalisées au logement porte aussi les conséquences de l'abattement forfaitaire de cinq euros décidé par le Gouvernement à l'été dernier. Cette mesure, initialement prise pour équilibrer le budget pour

Pour revenir à la mission, vous opérez un rebasage bienvenu concernant l'hébergement d'urgence et je ne peux, sur le programme 177, que partager votre priorité donnée à l'accès au logement, votre recherche d'une meilleure maîtrise des coûts et vos efforts pour restructurer le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion.

C'est désormais un fait : l'État se désengage complètement du financement des aides à la pierre, avec seulement 50 millions d'euros de crédits budgétaires inscrits. À la place, il est demandé aux bailleurs sociaux de financer davantage le Fonds Plus de crédits pour les aides à la pierre donc, en revanche, le budget de l'État fait son grand retour en tant que financeur de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH. Ainsi, 110 millions d'euros sont inscrits pour le programme Habiter mieux en 2018 et une enveloppe de 1,2 milliard d'euros est annoncée sur le quinquennat dans le cadre du Grand Plan d'investissement. Ces crédits viennent prendre le relais des crédits du programme Le budget de l'ANAH reste cependant soumis à l'aléa du cours des cessions de quotas carbone, mais paraît toutefois davantage sécurisé que par le passé, ce dont je ne peux que me réjouir. les crédits de la politique de la ville se trouvent globalement sanctuarisés. Les acteurs de cette politique publique ne sont toutefois pas rassurés, après la forte mesure de régulation budgétaire opérée au mois de juillet 2017 et ayant conduit à l'annulation de crédits remontés des territoires. Par ailleurs, le Gouvernement affiche de fortes ambitions en termes de rénovation urbaine, avec une enveloppe portée à 10 milliards d'euros pour le nouveau programme national de l'ANRU, paraît plutôt assurée à court terme, de même que le financement global du NPNRU- nous verrons avec les bailleurs sociaux -, plusieurs interrogations restent toutefois en suspens. Monsieur le ministre, comment comptez-vous couvrir l'impasse de trésorerie identifiée, non à court terme, mais sur le moyen ou le long terme ? Je Je terminerai mon propos en revenant sur l'article 52, qui, il faut bien l'avouer, a focalisé notre attention et nos échanges au cours des dernières semaines, et jusque tard dans la nuit ! À partir des mesures qui étaient proposées par le Gouvernement, nous avons mené, avec la commission des affaires économiques, mais aussi avec des sénateurs de divers groupes du Sénat, un important travail de concertation en vue d'un compromis. lors de l'examen de la première partie, à l'adoption d'un relèvement du taux réduit de TVA à 10 % pour les constructions et les travaux réalisés dans les logements sociaux, pour un rendement de 700 millions d'euros. Une première étape a été franchie.

la commission des finances a demandé l'examen de l'article 52 en priorité. Cela nous permettra ensuite d'examiner en connaissance de cause les crédits de la mission que la commission des finances vous proposera d'adopter en fonction de ce que nous aurons décidé sur cet article et dès lors que le Gouvernement aura présenté l'amendement annoncé lors de l'examen de l'article d'équilibre visant à inscrire 700 millions d'euros supplémentaires sur le programme 109, « Aide à l'accès au logement ». La parole

pouvez-vous nous indiquer à quelle logique répond ce changement ? Deuxièmement, les crédits consacrés aux contrats de ruralité diminuent et perdent en lisibilité. Ces contrats, nous les réclamions depuis longtemps, et j'avais moi-même proposé en 2016 dans un rapport d'information sur le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, le FNADT, qu'ils puissent être créés pour accompagner les stratégies de développement local des territoires ruraux.

Le projet de loi de finances pour 2018 conserve le dispositif, ce dont nous sommes satisfaits. Toutefois, en dehors des 44 millions d'euros de crédits de paiement prévus sur le programme 112 pour honorer les engagements de la seule année 2017, aucun crédit n'est réellement dédié aux nouveaux contrats de ruralité. Alors que, dans la loi de finances pour 2017,

Cela signifie donc qu'il n'y aura pas réellement de crédits disponibles pour financer de nouveaux contrats en 2018, sauf à consommer les crédits de droit commun inscrits sur la DSIL au détriment d'autres projets. pouvez-vous nous indiquer si de nouveaux contrats pourront être signés en 2018 et, si oui, avec quels crédits et pour quels montants ? Troisièmement, la prime à l'aménagement du territoire est une aide directe aux petites et moyennes entreprises qui vise à soutenir l'emploi dans les territoires les plus fragiles.

20 millions d'euros, c'est le minimum nécessaire pour accompagner les entreprises dans ces territoires, d'autant qu'une part importante de cette enveloppe sera consommée dans le cadre des engagements pris par l'État pour faciliter la reprise du site de Whirlpool à Amiens.

Pour ma part, je considère que cette agence devrait s'appuyer sur le CGET, dont l'expertise n'est plus à démontrer dans l'accompagnement des territoires. Monsieur le ministre, pourrez-vous nous en dire davantage sur la forme que pourra prendre cette instance ?

les équilibres trouvés pour ce site dont les enjeux dépassent largement le cadre régional. Je pense qu'il conviendrait, là aussi, de donner de la lisibilité aux nombreux acteurs locaux en les accompagnant mieux vers la sortie annoncée du dispositif.

monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les crédits des programmes 177, 109 et 135 diminuent pour atteindre 15,8 milliards d'euros pour 2018. Le Gouvernement a en effet décidé que la politique du logement participerait de façon importante à la baisse de la dépense publique. Ainsi, les crédits du programme 109 relatifs aux APL diminuent de 12 %. Le Gouvernement a absolument tenu à afficher une économie de 1,7 milliard d'euros sur les dépenses publiques, dont 1,5 milliard d'euros résultent de la création à l'article 52 d'une réduction de loyer de solidarité, la RLS, et à la baisse des APL qui en résulte. Certes, il faut faire des économies et la rigueur budgétaire s'impose à tous, mais cette mesure a été décidée brutalement et sans concertation, ni avec les bailleurs sociaux ni avec les élus. Le coût financier est important pour les bailleurs, bien au-delà de 1,5 milliard d'euros, car la RLS peut s'appliquer à des locataires « non APLisés », dont le Gouvernement ne peut chiffrer le nombre. De même, il faut ajouter les coûts de gestion supplémentaires qu'implique la RLS, ainsi que le coût du gel des loyers et le gel des barèmes de calcul des APL. Ces mesures coercitives auront nécessairement un impact en termes de construction et d'emploi dans les territoires ; elles fragiliseront un peu plus les collectivités territoriales par le biais des garanties d'emprunt en cas de défaillance des bailleurs sociaux. De plus, je reproche au Gouvernement de segmenter la réflexion. Or fragiliser l'un des maillons de la chaîne du logement menace l'ensemble d'un secteur qui marche. qui marche. Philippe Dallier, Sophie Primas, Valérie Létard, d'autres collègues et moi-même avons cherché une solution de compromis qui permette de réaliser des économies budgétaires et qui soit moins douloureuse pour les bailleurs sociaux. Ainsi, en complément de l'augmentation du taux de TVA estimée à 700 millions d'euros, j'ai proposé

Je ne nie pas la nécessité pour le secteur de devoir se restructurer. Il nous faudra, mes chers collègues, commencer à y travailler rapidement, afin d'être force de proposition lors de l'examen du projet de loi Logement. Sur le programme 135, les crédits diminuent également. En contradiction avec sa stratégie quinquennale censée créer un choc d'offres, l'État se désengage des aides à la construction, notamment des aides à la pierre. Ainsi, il ne contribuera au FNAP qu'à hauteur de 50 millions d'euros, alors qu'il oblige dans le même temps les bailleurs sociaux à augmenter leur contribution pour qu'elle atteigne 375 millions d'euros. Les aides aux maires bâtisseurs sont supprimées, le dispositif taux zéro, sont recentrés. Je salue en revanche l'engagement du Gouvernement à financer l'ANAH. Sur le programme 177, les crédits de la politique d'hébergement d'urgence augmentent de 12 %. Toutefois, nous pouvons légitimement nous interroger sur leur sous-budgétisation. En conclusion, la commission des affaires économiques s'en remet à la sagesse du Sénat sur les crédits des programmes 177, 109 et 135.

Rappelons que le Gouvernement s'est engagé à sanctuariser pendant le quinquennat les crédits dédiés à la politique de la ville et à ne pas procéder à des coups de rabot. Monsieur le ministre, nous veillerons au respect de ces deux engagements. Le Président de la République s'est également engagé à maintenir les dotations pour les communes en politique de la ville et a rappelé l'importance de « ramener le droit commun dans les quartiers, afin que chacun ait accès aux mêmes services ». Cela va dans le sens des préconisations que Valérie Létard et moi-même avons formulées, lors de notre mission d'information sur l'évaluation de la loi Lamy. S'agissant du NPNRU, le Gouvernement s'est engagé à porter le montant du programme à 10 milliards d'euros, dont un milliard d'euros seraient versés par l'État. Ainsi, l'État participera au financement du NPNRU à hauteur de 200 millions d'euros pendant le quinquennat, mais seulement de 15 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour 2018. Je considère que c'est un mauvais signal qui est envoyé pour

Comme Dominique Estrosi Sassone, je dénonce la brutalité de cette mesure. Les nouvelles marges de manoeuvre financières qui résultent de l'augmentation des crédits du NPNRU doivent permettre

ville. Le programme 147 consacre 106 millions d'euros au développement économique et à l'emploi. En outre, le Gouvernement a souhaité rétablir les emplois francs tout en en assouplissant les conditions. les conditions. Je m'interroge sur l'effet d'aubaine pour les entreprises, qui embaucheront des jeunes diplômés à moindres frais, alors même qu'il faudrait soutenir les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Pour ces derniers, les contrats aidés sont une bonne solution, contrairement à ce que nous pouvons entendre ; sur ce sujet, une évaluation serait bienvenue. En conclusion, la commission des affaires économiques s'en remet à la sagesse du Sénat pour le vote des crédits du programme 147 et émet un avis favorable sur l'adoption de l'article 58 , qui porte le montant du NPNRU à 10 milliards d'euros.

Ce programme est le réceptacle des insuffisances et des échecs de différentes politiques sociales et économiques, et chacun d'entre nous constate au quotidien combien la question du « sans-abrisme » a pris ces dernières années, et jusqu'à ces derniers jours, une acuité croissante. Face à la progression du nombre de sans-abri, les solutions sont notablement insuffisantes, alors que le droit à l'hébergement est inscrit dans le code de l'action sociale et des familles. Un chiffre, fourni par les annexes budgétaires, illustre cette insuffisance en 2017, seuls 21 % des demandes d'hébergement et 1 % des demandes de logement adressées aux services intégrés d'accueil et d'orientation ont pu être satisfaites. Au-delà des alternances politiques, les constats que je dresserai devant vous s'inscrivent malheureusement dans la continuité des exercices précédents. Comme chaque année, les crédits du programme 177 augmentent augmentent nettement. La progression était de 15 % l'année dernière, elle est de 12 % cette année, soit 212 millions d'euros supplémentaires par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Néanmoins, comme chaque année, les crédits qu'il nous est demandé de voter sont inférieurs à ceux qui auront réellement été consommés en 2017, compte tenu des dotations supplémentaires qui ont été nécessaires pour faire face à l'urgence.

sa volonté de ne pas recourir à des décrets d'avance en 2018 et tablerait par conséquent sur une baisse effective des dépenses du programme. Cette volonté n'est pas tenable, à moins de consentir à une augmentation drastique du nombre de personnes et de familles laissées à la rue. Il s'agit donc certainement d'un voeu pieux, qui accentuera les difficultés de trésorerie des opérateurs locaux. Cette insuffisance manifeste des crédits du programme 177 est à replacer dans le contexte de l'annonce par le Président de la République d'un plan quinquennal pour le logement d'abord. Il s'agit de recentrer les dispositifs d'hébergement sur la réponse à l'urgence et la mise en oeuvre du droit inconditionnel à l'hébergement et de rechercher une intégration rapide dans le logement, couplée à un accompagnement social renforcé. Ces orientations font consensus. Elles ne sont pour autant pas nouvelles. D'autres avant vous, monsieur le ministre, ont cherché à les mettre en oeuvre. Toutefois, la réussite d'un tel plan nécessiterait d'y consacrer des moyens nettement supérieurs le projet de loi de finances pour 2018. Favoriser l'accès direct au logement suppose par ailleurs de développer l'offre de logements très sociaux, et l'article 52 suscite un certain nombre d'inquiétudes quant à la capacité des bailleurs à réaliser les investissements nécessaires. La commission des affaires sociales considère donc que les crédits du programme 177 témoignent, comme chaque année, d'une sous-budgétisation et d'une insincérité préoccupante. S'agissant de l'adoption des crédits de l'ensemble de la mission, elle a émis un avis de sagesse. La parole

monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 17 juillet dernier, le Gouvernement s'est engagé dans une dynamique positive en faveur de la ruralité lors de la première Conférence nationale des territoires. Cinq mois plus tard, nous regrettons que les crédits dédiés à l'aménagement du territoire dans la mission examinée aujourd'hui ne traduisent pas fidèlement cette ambition.

Davantage qu'un simple ajustement technique, ce choix ne s'accompagne d'aucune garantie quant aux crédits d'engagement dédiés aux contrats de ruralité pour 2018. durable a donc exprimé de réelles inquiétudes quant à l'avenir de cet outil, pourtant apprécié par les acteurs locaux lors de sa première année de mise en service. Il s'agit en effet d'un instrument pertinent pour soutenir des projets transversaux de développement local qui contribue à la reconnaissance des problématiques spécifiques de la ruralité, à l'instar des contrats de ville pour certains territoires urbains. Nous avons par ailleurs relevé que plusieurs éléments constants du programme 112 continueront de diminuer en 2018. La commission a particulièrement souligné la nécessité de maintenir à un niveau suffisant

cette situation nous semble peu favorable à un véritable renforcement de l'ingénierie mise à disposition des collectivités, ingénierie que nous appelons de nos voeux. Nous avons toutefois salué l'effort décidé en faveur du développement des maisons de services au public, compte tenu de l'importante contribution de cette politique au maintien d'une offre de services publics de qualité et de proximité dans les territoires. La commission a par ailleurs relevé la création d'une nouvelle action au sein du programme 162, dédiée à la revitalisation du littoral occitan. Si les crédits demeurent très limités pour 2018,

Toutefois, son budget reste mineur en termes financiers. Il ne représente en effet que 3 % des crédits de la politique d'aménagement du territoire, soit 7,7 milliards d'euros en 2018.

Si nous n'investissons pas aujourd'hui dans un projet de cohésion globale de nos territoires, la France perdra demain son équilibre. À l'heure actuelle, deux programmes concourent à la politique de cohésion des territoires. Le programme 162, « Interventions territoriales de l'État » est le premier d'entre eux. Il comporte notamment les crédits du Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, le FACÉ.

encourage une révolution énergétique à grande vitesse, qu'il réduise parallèlement les crédits accordés à l'extension et au renforcement des réseaux de distribution d'électricité dans nos campagnes.

Cette diminution résulte essentiellement, cela a été dit par le rapporteur pour avis, du retrait du programme des contrats de ruralité. La force de la France, c'est pourtant la diversité de ses territoires. Les contrats de ruralité sont unanimement salués comme des outils pluriannuels de développement de notre territoire. Ainsi, 786 intercommunalités sont déjà engagées dans environ 500 contrats de cette nature, les objectifs étant d'améliorer l'accès aux soins, de revitaliser les centres-bourgs, ou encore d'accroître l'attractivité territoriale. Nous partageons l'inquiétude de nombre de nos collègues concernant l'isolement de ces contrats à l'extérieur du programme 112. 112. Quelques avancées notables au sein de ce même programme méritent cependant d'être saluées : le maintien de la prime d'aménagement du territoire, un des derniers régimes d'aide directe aux entreprises autorisés par l'Union européenne, le régime réformé

Toutes ces initiatives contribuent à recréer de l'emploi dans nos territoires et doivent être accompagnées par un maillage territorial resserré. C'est pourquoi mon groupe félicite le Gouvernement de sa décision d'augmenter de 3 millions d'euros les crédits accordés aux maisons de services au public.

cette seule mesure nous conduit à rejeter les crédits de cette mission. Pour finir, je dirai un mot, si vous me le permettez, sur la couverture numérique du territoire. La couverture mobile et internet de nos territoires est essentielle à leur attractivité. Le Gouvernement a fixé des objectifs ambitieux dans le courant du mois de septembre : bon haut débit pour tous dès 2020, très haut débit pour tous dès 2022 et couverture mobile de qualité généralisée d'ici à 2020. Nous soutenons ces objectifs, mais nous ne croyons pas que le niveau actuel des crédits de cette mission permettra de mettre en oeuvre de telles ambitions.

de la baisse drastique des APL, le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera contre les crédits de cette mission.

porter la mission « Cohésion des territoires », laquelle subit la plus forte baisse de crédits au sein du projet de loi de finances pour 2018, et mener de front la réforme du logement dont nous avons tant besoin, la situation urgente dans laquelle se trouvent 4 millions de nos concitoyens mal logés, n'est pas un exercice aisé. Je le conçois volontiers, monsieur le ministre. Cette tâche est d'autant plus complexe et sensible que nous touchons en l'espèce à l'un des besoins les plus fondamentaux : le droit de chacun de vivre dignement dans un logement décent.

Le programme 109, « Aide à l'accès au logement » concentre 82 % des crédits de la mission pour un montant de 13,6 milliards d'euros.

Toutefois, nous aurions souhaité que la baisse des aides au logement prévue à l'article 52 intervienne de manière plus équitable, dans le cadre d'une réforme globale, indépendamment des considérations purement budgétaires, puisque cette mesure permet de réaliser une économie de 1,5 milliard d'euros. Si j'entends l'argument selon lequel les APL auraient un effet inflationniste, bien que celui-ci soit difficile à évaluer avec exactitude, leur baisse prévue dans le présent projet de loi aura avant tout des effets sur le logement social, c'est-à-dire le secteur où les loyers sont contrôlés. Or c'est dans le secteur privé que les loyers demeurent excessifs. Je rappelle en outre que la moitié des personnes vivant sous le seuil de pauvreté réside dans le parc privé et paie des loyers de 40 % à 50 % plus élevés, comme l'a souligné la Cour des comptes en février dernier. J'en viens aux effets de l'article 52 sur la capacité de financement des bailleurs sociaux, dont la situation financière globale est certes confortable. Le problème est que cet article frappe indistinctement leur capacité d'autofinancement, alors qu'ils ne font pas tous partie des structures ayant rentabilisé leur patrimoine sans pour autant avoir investi dans la construction ou l'amélioration du parc social. Frappés par la réduction de loyer de solidarité, ils devront par ailleurs contribuer au doublement du nouveau programme national de renouvellement urbain. Nous espérons que le dispositif de péréquation et le mouvement de restructuration permettront de résoudre ces difficultés. Le Sénat devrait parvenir à proposer une solution intermédiaire, après l'adoption en première partie de la hausse de la TVA sur la construction et la réhabilitation des logements sociaux. D'autres leviers seront bienvenus. Je pense à la prise en compte des revenus de l'année en cours pour les bénéficiaires des APL, laquelle devrait s'appliquer en 2019, ou encore à la réflexion sur une meilleure application du supplément de loyer de solidarité. Au-delà de la polémique, il est essentiel de s'interroger sur le modèle du logement social, qui devrait être réservé en priorité aux ménages modestes et défavorisés. Or le taux de rotation reste faible, ce qui exclut de fait ces derniers. Il convient, en parallèle, d'accélérer le développement de l'offre de logements à des prix accessibles dans les zones tendues pour mettre fin au cercle vicieux dans lequel la dépense publique ne cesse d'augmenter pour répondre imparfaitement aux dysfonctionnements du marché immobilier. L'accession à la propriété doit faire l'objet d'une plus grande attention. Il faut faire en sorte que plus de locataires deviennent propriétaires au lieu de concentrer

leur vie. Les ménages modestes doivent pouvoir acquérir leur logement. D'après le rapport de la commission des finances, le taux de propriétaires parmi les 25-44 ans a diminué de 53 diminué de 53 % entre 1973 et 2013, alors qu'il a augmenté dans les mêmes proportions chez les ménages aisés. Le groupe du RDSE soutiendra ainsi le rétablissement des APL-accession. Par ailleurs, j'évoquerai brièvement, en raison du peu de temps qui m'est imparti pour évoquer une si vaste mission, l'augmentation des crédits relatifs à l'hébergement d'urgence, programme qui était frappé par une sous-budgétisation chronique. Je tiens donc à saluer l'objectif très ambitieux du Gouvernement qui vise à ce que plus personne ne dorme dans la rue. Monsieur le ministre, je sais avec quelle fermeté vous défendez l'égalité des territoires, alors que de fortes disparités demeurent. Or, lorsque les territoires sont isolés, la cohésion prend une tout autre dimension : l'abandon n'est pas qu'un simple sentiment. Tous les territoires doivent bénéficier de cette solidarité, ceux qui, comme Saint-Martin, la Guyane

ministre, que nous avons exprimées n'altèrent en rien l'admiration et le respect que nous vous portons et ne remettent nullement en cause la confiance que nous avons en vos qualités d'écoute, de discernement en votre pouvoir de persuasion. Ainsi, dans sa grande majorité, le groupe du RDSE porte un regard bienveillant sur le travail de concertation que vous engagez et fera confiance à votre sens de l'équité.

Cette mission et ses articles rattachés ont suscité, je l'ai entendu, de nombreuses interrogations, l'article 52 ayant été au centre de l'attention médiatique et parlementaire. En ces temps de discussion et de négociation, le Gouvernement a fait preuve d'ouverture et d'écoute, tout en présentant une ligne claire et exigeante sur ce sujet à la fois technique et important pour le quotidien des Français. Quelles sont les bases de ce débat ?

la qualité et la stabilité du logement. Au total, la France compte 4 millions de mal-logés ! Cette réalité doit nous pousser à agir. C'est ce chantier qu'entame aujourd'hui le Gouvernement. il faut bien avoir en tête la volonté du Gouvernement que partage la majorité présidentielle : elle est bien de défendre le modèle du logement social français. Et pour ce faire, il faut améliorer ce modèle, le rendre plus efficace pour les locataires et pour les organismes. Il y a beaucoup à faire. Je pense que nous pouvons être fiers de la réflexion engagée par le Gouvernement.

Tout le monde aura noté les avancées lors du débat parlementaire : une stabilisation du taux du livret A qui entraînera un gain de 700 millions d'euros, mais aussi des facilités de prêts. Au total, c'est un paquet financier inédit pour le logement social, qui ne bénéficie pas des taux extrêmement faibles que l'on connaît.

mais les organismes ont mis en avant leur préférence pour une hausse du taux de la TVA sur la construction et la rénovation. Une augmentation de ce taux de 5,5 % à 10 % rapporterait 700 millions d'euros. Le Sénat a voté en faveur de cette hausse de TVA. C'est un premier pas, mais il faut aller jusqu'au bout et ne pas en rester à cette demi-mesure.

et au secrétaire d'État ici présents. Ils ont mené cette concertation depuis l'été, en rencontrant les bailleurs sociaux. Ils sont largement responsables de ce compromis, qui devrait aboutir dans les jours qui viennent. Pour toutes ces raisons,

Je pourrais citer plusieurs indicateurs assez parlants, comme l'ancienneté moyenne des locataires du parc social, qui est de treize ans contre sept ans dans le parc privé, ou encore l'insuffisance de petits logements, autrement dit l'inadéquation entre la demande et l'offre, et enfin, une liste d'attente sur laquelle figurent près de 1,5 million de demandeurs.

Ces deux décisions reflètent bien les deux volets de la politique du logement de ce gouvernement : une externalisation de ses financements et une politique au rabot guidée par l'objectif de réduire les dépenses publiques. en quelque sorte, de répondre à la crise du logement, qui pourtant s'aggrave. La France compte ainsi plus de 4 millions de mal-logés et plus de 15 millions de personnes souffrant à des degrés divers du mal-logement. En outre, 1,9 million de personnes sont dans l'attente d'un logement social. vivant ces situations personnelles douloureuses, le coup de rabot de cinq euros sera extrêmement difficile à assumer. Nous soutenons donc le collectif Vive l'APL, qui fédère tous les opposants à cette décision inique. Loin d'être révolutionnaire, ce budget pousse la logique de désengagement à son paroxysme et risque d'accroître les difficultés sociales en portant atteinte au modèle économique du logement social dans notre pays,

abordables. Le FNAP, dont nous avons dit à plusieurs reprises qu'il serait l'outil du désengagement de l'État, est dorénavant financé à titre principal par les bailleurs sociaux, à hauteur de 86 % de son budget. Ce sont donc les locataires qui le financent. La boucle est bouclée

Les bailleurs sont sommés de financer non seulement le FNAP, mais aussi le plan de rénovation urbaine à hauteur de 2 milliards d'euros supplémentaires, selon les dernières annonces concernant le doublement du NPNRU.

la baisse des loyers dans le secteur public concomitante à la baisse des APL à hauteur de 1,5 milliard d'euros, comme le prévoit l'article 52.

Toutes ces mesures concourent à faire des bailleurs, du 1 % logement et des collectivités les principaux contributeurs au financement du logement public. Contrairement

Ces mesures risquent également de menacer l'équilibre de certaines opérations, voire de conduire à la faillite un certain nombre de bailleurs, sans parler des collectivités qui en sont aujourd'hui les garantes.

locatifs. La cohésion territoriale ne passant pas uniquement par une réforme du logement, nous devons concevoir et promouvoir un développement qui ne stigmatise pas les territoires à faible démographie. Il faut au contraire en faire des exemples en matière de développement durable, de cohésion sociale, de vivre ensemble, de culture et d'éducation. Le développement équilibré de nos territoires ne se fera pas sans une complémentarité entre l'urbain et le rural, et ce sans hiérarchie ni condescendance. La ruralité La ruralité est un socle de savoir-faire, de savoir-être et d'initiatives porteuses. Ainsi, le renforcement des coopérations entre tous les territoires sera le fondement d'un futur favorisant la transition écologique, économique et sociale.

la mission « Cohésion des territoires » rassemble désormais les programmes précédemment rattachés aux missions « Égalité des territoires et logement » et « Politique des territoires ». Pour cette mission, qui comporte six programmes,

Le Gouvernement s'est toutefois engagé à porter les crédits du NPNRU de 5 milliards d'euros à 10 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur la durée du programme. Cet engagement est inscrit à l'article 52 . Nous y sommes favorables.

Toutefois, certaines interrogations demeurent. Ainsi, si le présent projet de budget acte le retour de l'État dans le financement du renouvellement urbain aux côtés d'Action Logement et des bailleurs sociaux, ce retour reste balbutiant. L'État participera au financement du NPNRU à hauteur de 1 milliard d'euros sur la durée du programme, dont 200 millions d'euros pendant le quinquennat. Or comment compte-t-il tenir cet engagement alors que, pour 2018, seuls 15 millions d'euros sont inscrits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement ? difficile de ne pas se montrer sceptique quant à la réalisation des engagements de l'État. Il ne faut en effet pas oublier que, cet été, le décret d'avance du 27 juillet 2017 a annulé les 100 millions d'euros inscrits en autorisations d'engagement ainsi que les 15 millions d'euros de crédits de paiement inscrits dans le budget pour le NPNRU- soit l'intégralité des budgets pour l'année 2017 ! Au total, ce sont 130,4 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 46,5 millions d'euros de crédits de paiement qui ont été annulés, ce qui est considérable. Par ailleurs, si l'article 52 porte le NPNRU à 10 milliards d'euros, se pose encore la question du financement de cette augmentation. Comment l'État va-t-il trouver les 4 milliards d'euros qui manquent pour financer le NPNRU ? ? Ne l'oublions pas non plus, en parallèle à ces mesures, l'article 52 du projet de loi de finances pour 2018 impose, en contrepartie de la baisse des APL dans le logement social, une réduction des loyers de solidarité finalement étalée sur trois ans. Pour l'année 2018, la baisse des loyers correspondra à une perte de pas moins de 822 millions d'euros, qui devra être absorbée par les 254 offices publics de l'habitat qui détiennent 2,5 millions de logements. À cela s'ajoutent plusieurs autres mesures qui vont peser principalement sur les bailleurs comme la hausse de leur participation au Fonds national des aides à la pierre. Ces mesures, qui interviennent en pleine négociation du futur NPNRU 2018-2024, vont directement impacter la capacité d'autofinancement des organismes d'HLM, et nécessairement fragiliser la politique locale en faveur du logement social. C'est l'ensemble des projets de rénovation urbaine déjà engagés ou simplement prévus qui pourraient être remis en cause. Un accord a été trouvé le 21 novembre dernier avec Action Logement, qui financera 2 milliards d'euros supplémentaires. Le financement du NPNRU sur l'ensemble du quinquennat n'est cependant pas encore bouclé. Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'être inquiets sur l'avenir du logement social et la concrétisation des contrats de ville qui ont été signés et qui préfigurent la conclusion des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain. La brutalité de l'ensemble de ces mesures et l'absence de concertation laissent à penser que la seule ligne directrice du Gouvernement est la réalisation de 1,7 milliard d'euros d'économies, et ce sans véritable politique du logement et de la mixité sociale.

au risque de mettre à bas le monde du logement social, mais aussi avec son lot de conséquences sur les collectivités, avant même l'examen de la loi qui doit arriver au printemps et dont l'objet est d'établir une véritable réforme du logement

? La mesure budgétaire proposée par l'État, si elle peut se comprendre sur le fond, n'est pas acceptable quant à la méthode, trop brutale et sans concertation. Où sont les collectivités dans ce débat ?

ambitions s'inscrivent dans une logique de justice comme la volonté de favoriser l'accession à la propriété dans le cadre d'un parcours résidentiel efficace, comme la volonté d'accélérer la rénovation ou de relancer la construction de logements.

que vous prétendez poursuivre, car force est de constater que les choix budgétaires du Gouvernement montrent que vous aggraverez la situation du logement et des moins aisés. Mesurez les effets de cette baisse de 1,5 milliard d'euros supportés par les bailleurs sociaux. Les coupes opérées sont bien des coupes claires et non des coupes sombres, comme l'aurait précisé Jean d'Ormesson. Par cette décision, vous obérez d'une manière irréversible et inacceptable le modèle économique du logement social avec des effets dévastateurs sur la construction de logements, sur la réhabilitation des logements, et après avoir organisé le plus grand plan social par la remise en cause des contrats aidés, vous continuez votre forfait sur l'emploi dans ce secteur, avec plus de 140 000 emplois concernés. Cette perte de recettes de 1,5 milliard d'euros, c'est 70 % de la capacité d'investissement des organismes d'HLM, c'est 54 000 logements qui ne seront pas construits, c'est plus de 100 000 logements qui ne seront pas réhabilités.

Dans le cadre d'une conférence de consensus, nous ne sommes d'ailleurs pas opposés à une évolution de ce modèle. Et le Sénat, dans sa grande sagesse, sur toutes ses travées, avait accepté la recherche d'un compromis qui, notamment, prenait la forme d'une augmentation de la TVA applicable aux opérations réalisées dans le logement social, un compromis qui tenait compte des revendications de l'Union sociale pour l'habitat, un compromis qui intégrait même votre cadre budgétaire de 1,5 milliard d'euros, mais qui préservait le modèle économique du logement social en France. Ce compromis, vous tenterez de le balayer dans quelques instants en faisant porter vos réductions de crédits par une baisse des loyers irréversible de 800 millions d'euros sur la RLS, comme l'indique l'amendement que vous Que reste-t-il d'une stratégie politique lorsqu'elle est animée par une logique budgétaire ? Quelle est votre vision pour permettre à tous de vivre dans un logement décent et abordable ? Vous diminuez les aides à la personne, avec la baisse des APL, la suppression de l'APL-accession, et, dans le même temps, les aides à la pierre, avec le désengagement de l'État à hauteur de 75 % du Fonds national aux aides à la pierre, avec la suppression de l'aide aux maires bâtisseurs qui entraînera inévitablement un frein à la construction de logement. Peut-être avez-vous une vision ? Peut-être, après la destruction de ce modèle, souhaitez-vous lui substituer un autre système ? Dans ce cas-là, dites-le-nous, dites-le aux bailleurs, dites-le aux professionnels de la construction et aux Français en général. Vous leur devez de la transparence. À l'écoute de tous les acteurs du secteur du logement, nous sommes face à vous pour porter des propositions afin de lui redonner de la justice et de la solidarité, pour rendre une cohérence économique à la politique du logement présentée dans cette seconde partie du projet de loi de finances. Par amendement, le groupe socialiste et républicain défendra la suppression de l'article 52, le rétablissement de l'aide aux maires bâtisseurs et l'augmentation de la contribution de l'État à l'aide à la pierre pour maintenir le niveau d'engagement de 2017. Face à vous, nous prenons notre place de défenseurs de ce modèle qui protège les ménages les plus modestes, grâce à un modèle économique et social qui les a notamment protégés lors de la crise de 2008. Permettez-moi une dernière

Car, malheureusement, l'instauration d'un ministère spécifique et la volonté de créer une agence des territoires ne s'accompagnent pas des crédits nécessaires. Si quelques bonnes dispositions figurent dans votre budget, le sentiment général est proche de la déception. La mise en place de la conférence des territoires avait suscité des attentes de la part des élus et des citoyens qu'ils représentent. Je rappelle que le Président de la République avait, en juillet, indiqué : « Ce que demande la ruralité [ ...], c'est d'avoir les mêmes chances de réussir. La création d'une agence des territoires, telle l'ANRU, devait être porteuse de ce souffle nouveau. Mais au regard des chiffres, notamment la forte baisse des crédits dédiés au Commissariat Au-delà des chiffres, il y a bien un sentiment d'abandon, je dirai même de défiance, de la part des ruraux. Lors du dernier congrès des maires de France, ce sentiment est remonté jusqu'à vous. En effet, les motifs de préoccupation sont nombreux : fin de la dotation d'action parlementaire, suppression de 209 millions d'euros de crédits consacrés à la DETR, réforme de la taxe d'habitation, objectif de baisse de 13 milliards d'euros sur les dotations de l'État aux collectivités, absence de réforme de ces dotations, qui pénalise les communes rurales, réduction du nombre d'élus locaux et de parlementaires. Bref, la ruralité est inquiète, et votre budget en matière de cohésion des territoires ne pourra pas la rassurer. Mais revenons au projet de loi de finances, plus précisément aux programmes 162 et 112. D'abord, j'aimerais indiquer que les changements de périmètre de la mission n'ont pas facilité la compréhension de votre politique. de l'État, le PITE, les crédits sont en légère hausse. Je ne peux que m'en réjouir, car cela touche directement ma région et mon département avec le plan Littoral 21. L'État se grandit d'avoir une continuité sur des projets environnementaux d'envergure. Nous serons néanmoins vigilants dans l'application réelle de vos ambitions. En revanche, sur l'autre programme, le 112, celui qui concerne directement la politique d'aménagement du territoire, on assiste à un désengagement. Les crédits sont en net retrait par rapport aux budgets antérieurs, déjà faiblement dotés. En décidant de réduire de 58 % les autorisations d'engagement pour ce programme, vous désincarnez toute une politique qui a fait ses preuves. Au sujet des contrats de ruralité, les projets à venir ne trouveront pas les crédits nécessaires.

Je le regrette, car au-delà de la déception des élus, des projets d'avenir visaient des territoires en difficultés. La ruralité peut être une terre de croissance et de développement, si on lui en donne les moyens. Mais ceux-ci manquent terriblement à votre budget. Le Gouvernement aura beau indiquer que ces contrats seront financés autrement, cette confusion ne grandit pas vos ambitions en matière territoriale. À cela s'ajoute la division par deux, depuis cinq ans, de la dépense fiscale consacrée aux ZRR et le flou persistant pour les communes rurales intégrées à de grands EPCI. Dans mon département, une bonne partie des communes cévenoles sont rattachées à la communauté d'agglomération d'Alès qui compte 73 communes depuis les fusions imposées par la loi NOTRe. Si elles perdent le bénéfice du classement en ZRR, ces communes, dont certaines sont en grande souffrance, verraient leur attractivité réduite. Bien qu'il ne relève pas de cette mission, j'aurais pu aussi parler du Fonds d'intervention pour les La présence de services à la personne, comme celle des services publics, est la condition du développement de la ruralité. Ainsi, je me réjouis que vous décidiez d'accroître légèrement les financements des maisons de services au public. Néanmoins, cette évolution ne doit pas être le bras armé de la dévitalisation des secrétariats de mairie, qui sont la première interface, et souvent la seule, pour nos concitoyens. Absolument ! La question du maintien des services publics en zone rurale est un vrai sujet, et nous serons vigilants. monsieur le secrétaire d'État, mis à part quelques évolutions positives, la mission n'a, dans son ensemble, pas de dynamique ni même de sens. C'est profondément décevant.

Plus largement, je regrette que l'État ne soit plus stratège et n'ait plus aucune ambition en matière d'aménagement du territoire en zone rurale. En effet, au-delà de la baisse des crédits, il faut souligner l'absence de vision et de grands projets publics ruraux.

les crédits consacrés à l'aménagement du territoire au sein de la mission « Cohésion des territoires » sont, pour 2018, en légère augmentation en crédits de paiement- de 2 % exactement

Pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, cette division par deux des crédits pour les années à venir n'est évidemment pas un bon signe ; nous en sommes extrêmement inquiets. peut trouver des explications à cette situation, en particulier le transfert des crédits des contrats de ruralité vers un autre programme. Toutefois, cette évolution de périmètre ne comporte aucune garantie sur le maintien d'une enveloppe dédiée aux contrats de ruralité pour les années à venir dans le cadre de cette autre mission. De nombreux territoires se sont organisés pour faire appel à cet instrument, mis en place voilà à peine plus d'un an. Je le rappelle, près de 500 contrats sont conclus ou en cours de négociation n'est pas acceptable, car les élus ont besoin d'une stabilité du cadre et des règles qui leur sont applicables. Mon groupe est d'autant plus sensible à cette question qu'il a été à l'origine de la réflexion sur ces contrats, inspirés des contrats de ville, mais adaptés au monde rural.

ministre, monsieur le secrétaire d'État, rejoignent celles qui ont été exprimées par notre excellent rapporteur Louis-Jean de Nicolaÿ, que je salue. Il s'agit d'abord de la baisse de moitié de ce qui restait de la prime d'aménagement du territoire, heureusement légèrement amoindrie lors du débat à l'Assemblée nationale. Il s'agit ensuite de l'avenir très incertain de la dynamique des pôles de compétitivité dont la troisième phase doit s'achever en 2018. Nous aimerions savoir, monsieur le ministre, si vous allez poursuivre cette politique qui a eu un rôle structurant pour le développement d'écosystèmes régionaux, et selon quelles priorités. Il s'agit enfin de la politique des centres-bourgs, un sujet majeur pour les territoires et pour le Sénat, et sur lequel un groupe de travail piloté par Rémy Pointereau et Martial Bourquin doit réfléchir au cours des prochains mois. Mais, nous le savons tous, il ne peut y avoir de politique d'aménagement du territoire digne de ce nom si les deux priorités de nos concitoyens et des élus locaux sur les territoires ne sont pas mieux traitées : la couverture numérique et l'accès aux soins. Sur l'accès au numérique par les réseaux fixes et mobiles, qu'il s'agisse du haut débit fixe, du très haut débit fixe ou de la téléphonie mobile, le Gouvernement a fixé des objectifs. Nous les partageons.

Sur l'accès aux soins, il devient lassant d'entendre sans arrêt les gouvernants successifs faire un constat et annoncer des plans

messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, rétrospectivement et hors PNRU, la remarquable stabilité des crédits du programme 147 atteste que le Gouvernement inscrit son action dans le prolongement de la refondation opérée en 2014 par la loi Lamy et à la citoyenneté. Pour l'ensemble des acteurs de la politique de la ville, l'efficience doit être le maître mot de l'action publique dans les quartiers, au service des habitants et avec eux, dans la conception de l'agenda qui les concerne directement et dans l'évaluation, avec eux toujours, de l'action menée. Les acteurs de la politique de la ville ont besoin de visibilité et de garanties. Le chef de l'État a pris des engagements à Tourcoing. Nous serons vigilants sur leur respect. Dans le peu de temps qui m'est imparti, je voudrais aborder les conditions d'engagement du NPNRU dont les crédits d'engagement ont été portés à 10 milliards d'euros sur la durée du programme 2014-2024. Au-delà de la participation de l'ANRU au financement de ces programmes, la capacité contributive des collectivités locales interroge, tant leur contribution forte au rétablissement des comptes publics réduit incontestablement leur niveau d'intervention. Le modèle national du logement social étant également mis à mal par les mesures de baisse des loyers et des APL, les organismes d'HLM s'interrogent aussi sur leur propre engagement dans la durée. Dans ce contexte de difficulté et d'incertitude, les 200 millions d'euros de crédits de paiement prévus sur le quinquennat apparaissent comme insuffisants pour créer auprès des autres partenaires l'effet de levier nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous proposons un amendement portant à 100 millions d'euros les crédits de paiement pour 2018 de l'action n° 04, Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie, du programme 147. En conséquence, trois mesures apparaissent indispensables pour que le NPNRU s'engage dans un cadre partenarial efficace et durable : d'abord, la révision du calcul de la participation de l'ANRU, le fameux, pour tenir compte objectivement de la situation descollectivitésqui veulent s'engager ensuite, la redéfinition des règles de participation des bailleurs sociaux, notamment pour les démolitions ; enfin, dernier point lié aux deux autres, le relèvement de la participation financière de l'ANRU qui devrait se situer au même niveau que celle d'Action Logement. L'efficience de la politique de la ville sera aussi fonction de la pertinence des stratégies territoriales développées en matière de logement et de peuplement. Dans un contexte sociologique et culturel aujourd'hui très différent, et souvent plus compliqué, ne répétons pas les erreurs d'hier que nous tentons aujourd'hui de corriger avec des moyens somme toute considérables. Concrètement, les ménages les plus pauvres ne doivent pas être systématiquement orientés vers les quartiers engagés dans un programme de renouvellement urbain. La politique de peuplement doit être définie à l'échelle de territoires d'habitat dépassant largement le périmètre des quartiers et des villes abritant ces quartiers. C'est à ce prix que la mixité sociale pourra prendre une dimension spatiale et géographique adaptée aux enjeux de long terme. Tout à fait ! Les politiques du logement et de la ville doivent donc être liées par la problématique du peuplement. Pour ces raisons, nous pensons que le plan gouvernemental Logement d'abord doit aussi être mis en oeuvre dans le cadre d'une stratégie de peuplement globale et cohérente avec celle des quartiers. Une part des crédits de l'action n° 03, Stratégie, ressources et évaluation, doit donc être consacrée à la définition et à la mise en oeuvre, toujours propre à chaque territoire, de stratégies de peuplement marquées du sceau des valeurs de la République. Pour conclure, compte tenu des incertitudes relatives aux capacités contributives effectives des partenaires financeurs et à la pertinence des stratégies de peuplement, nous émettrons un avis de sagesse sur les crédits de cette mission.

En septembre, le Gouvernement a annoncé un choc de l'offre de logements. Nous sommes évidemment prêts à soutenir cet objectif. Mais les mesures que vous nous présentez, si elles ne sont pas amendées dans la loi de finances, vont provoquer un contre-choc Oui, nous avons besoin de construire 450 000 logements environ par an pour répondre aux problématiques de la natalité, de la décohabitation des couples et de l'allongement de l'espérance de vie. Contrairement à ce que j'ai entendu dans votre bouche et dans celle du Président de la République quand il est venu à Lille, nous avons déjà élaboré des projets qui marchent, comme dirait Mao Tsé-Toung,

quadruplement de l'accession sociale à la propriété, le doublement du financement social du logement, l'augmentation de 50 % de l'offre de construction, avec, au final, 5 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires par rapport aux dépenses, y compris les APL, et avec une martingale gagnante

C'est la faille de votre programme, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, au-delà des réductions purement comptables sur lesquelles je ne reviens pas : vous ne faites pas confiance aux acteurs du logement, en particulier aux bailleurs sociaux. À ce titre,

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, après ce concert de louanges, j'ai toujours autant de plaisir à m'exprimer devant le Sénat de la République

politiques, depuis 1997, ont participé aux gouvernements successifs de la République, y compris le groupe que j'ai représenté. Voilà la réalité. Nous avons donc, les uns et les autres, depuis vingt ans, assumé des politiques qui ont aggravé les déséquilibres territoriaux. Voilà le constat. Je ne dis pas que, par un coup de baguette magique, nous allons révolutionner les choses et que le bonheur va aussitôt inonder nos territoires. Je dis simplement que cette situation ne remonte pas au mois de mai 2017.

Au titre de ce budget, que j'assume avec les difficultés qui en découlent, nous avons pris un certain nombre de mesures qui permettront d'avancer de manière positive dans les années qui viennent.

Elle regroupe pour la première fois les soutiens financiers de l'État à la politique d'aménagement du territoire, à la politique de la ville et au logement. C'est vrai, à la demande du Président de la République, nous avons engagé une réforme profonde de la politique du logement dans notre pays. Oui, certaines décisions sont d'ordre budgétaire : je les assume.

elle doit être mise en cohérence avec la réforme financière des aides au logement que nous avons engagée. Nous sommes venus devant vous avec un texte voté par l'Assemblée nationale

des solutions et initiatives issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Selon nous, cette plateforme nationale pourrait être dénommée « agence des solutions locales ». Il s'agissait d'évaluer l'opportunité de créer une telle structure pour faciliter le soutien particulier des acteurs économiques, des collectivités territoriales et des services de l'État autour de ces initiatives : à terme, l'enjeu est de développer ces dernières à plus grande échelle. Nous voyons mal en quoi la rédaction d'un rapport crée une charge nouvelle pour l'État, sauf à considérer le travail de l'administration comme tel. Cette application erronée de l'irrecevabilité financière prive les parlementaires que nous sommes de leur droit d'amendement, qui est pourtant inaliénable : à l'évidence, on voudrait faire de nos assemblées de simples chambres d'enregistrement

La fracture territoriale et la fracture sociale s'aggravent chaque jour. Elles portent un coup terrible au pacte républicain et ouvrent la voie à de terribles maux. Les difficultés concentrées dans ces quartiers sont nombreuses

élus de tous bords politiques, animés encore d'espoir et de pragmatisme, se sont réunis le 16 octobre dernier pour lancer cet appel. Ensemble, ils ont construit une plateforme regroupant dix mesures d'urgence à prendre immédiatement dans ce budget pour

La commission des finances a mis en place une cellule spécifiquement dédiée à cette question. Les décisions ne sont jamais prises à la légère : les amendements sont analysés par les administrateurs de la commission, puis soumis au président de la commission des finances. Lorsqu'ils sont déclarés irrecevables, c'est toujours pour une bonne raison

C'est forcément pour l'une de ces raisons- croyez-moi, je doute beaucoup que ce soit à tort ! -que vos amendements ont été déclarés irrecevables.

Pour justifier cette mesure, le Gouvernement invoque une hausse exponentielle des sommes consacrées au financement des APL, à hauteur de 18 milliards d'euros, qu'il faudrait d'urgence contenir. Il est vrai que, depuis les années 1970, les pouvoirs publics ont fait le choix d'attribuer des aides au logement plutôt que des aides à la pierre, nous conduisant à la situation que nous connaissons aujourd'hui trop peu de logements pour absorber la demande sociale et, donc, des loyers élevés, le marché étant particulièrement déséquilibré. La démarche de ce gouvernement ne s'inscrit pas dans cette problématique, puisque la baisse des APL ne se conjugue pas avec une hausse des aides à la pierre. La justification politique est En effet, comment ne pas voir que la hausse des crédits des APL est imputable non pas aux bailleurs publics, dont les loyers sont réglementés, mais à la hausse des loyers dans le secteur privé, les aides au logement étant alignées sur le niveau de loyers Pour cette raison, nous sommes inquiets de la remise en cause de l'encadrement des loyers, qui risque d'entraîner de fait une dépense publique supplémentaire en matière d'APL, une dépense importante, faute de régulation des pouvoirs publics. Parlons également du niveau réel de contribution des entreprises au 1 % logement qui finance ce fonds.

la hausse de crédits est imputable non pas aux politiques du logement, mais bien à la pauvreté qui gagne du terrain dans notre pays et à la précarité qui gangrène notre société. Ce n'est donc pas en baissant les APL que nous réglerons cette situation ; c'est en s'attaquant directement aux causes, plutôt qu'aux conséquences. Renforcer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, c'est agir efficacement pour la baisse du niveau de financement public consacré aux APL, puisque cette aide est fonction des ressources du ménage. Nous pensons donc que nous nous engageons dans un mauvais débat avec cet article 52 tel qu'il est rédigé. Nous avons déposé un certain nombre d'amendements pour limiter

le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous parlerai de mon territoire, l'Aisne. Avec une production annuelle de 230 logements, 90 logements démolis et 50 logements vendus aux locataires, l'office d'HLM de l'Aisne et de Laon, que je présidais encore il y a quelques semaines, est un acteur local indispensable au territoire : 200 logements réhabilités thermiquement par an, 50 millions d'euros d'investissements annuels, plus de 500 emplois non délocalisables. Or la réforme des APL va transformer un office d'HLM sain en un office d'HLM déficitaire. En ce qui concerne mon office, plus de 6 millions d'euros par an sont en jeu. Le voilà déficitaire et rendu par vos mesures, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire De plus, cette réforme va mettre en difficulté les collectivités qui en sont les garantes. Ainsi, les offices qui ont joué le jeu en investissant régulièrement pour améliorer la qualité de l'habitat, mais qui ne disposent pas d'une trésorerie illimitée, vont subir la réduction de loyer qui leur sera imposée.

et/ou, souvent, d'un impôt sur la plus-value plus faible, la plus-value étant particulièrement exorbitante dans ces territoires. Pour lutter contre cette rétention foncière et créer un « choc d'offres », la loi prévoira, comme vous l'avez rappelé, que les vendeurs bénéficieront, pendant une période transitoire de trois ans, d'un abattement de 100 % pour la vente vente d'un terrain à bâtir situé en zone tendue, en vue de construire un logement social ; de 85 % pour la vente d'un terrain à bâtir situé en zone tendue, en vue de construire un logement intermédiaire ; et de 70 % pour pour la vente d'un terrain à bâtir situé en zone tendue, en vue de construire un logement dans le secteur libre. Cette disposition va, de toute évidence, monsieur le ministre, l'activité immobilière et la construction de logements sociaux ; nous y sommes, pour notre part, très favorables. Cependant, la loi ALUR, la loi

Au final, il préfère souvent ne pas vendre. Monsieur le ministre, ma question est la suivante : peut-on espérer de manière claire l'extension à tous les DOM et à La Réunion de la mesure très attendue du classement en zone tendue et du bénéfice de l'abattement précité pour la vente des terrains destinés au logement social et au

monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis défavorable à l'adoption de l'article 52, qui constituerait une bien mauvaise surprise, une bien mauvaise nouvelle pour les ménages modestes qui souhaitent devenir propriétaires, en ce qu'il prévoit la suppression du dispositif APL-accession. Or ce dispositif leur permet de devenir propriétaires de leur résidence principale tout en percevant des aides personnalisées au logement, au travers de deux types de crédit, le prêt d'accession sociale, le PAS, et le prêt conventionné. Les deux prêts permettent de financer jusqu'à 100 % du montant de l'opération envisagée- achat dans le neuf ou dans l'ancien, construction de maison -, pour une durée pouvant aller jusqu'à trente-cinq ans dans certains cas. En outre, cette aide est directement versée à la banque prêteuse et vient donc réduire la mensualité de crédit payée par l'emprunteur- jusqu'à 50 % dans certains cas la prenant en compte dans leurs plans de financement. Cela permet à des ménages dont l'endettement aurait été trop élevé sans aide de devenir propriétaires. Ainsi, on le voit bien, l'APL-accession est l'une des aides les plus efficaces. De plus, l'APL-accession, qui représente une part très réduite des APL, à savoir 5 % du budget total des allocations logement, soit 834 millions d'euros, a bénéficié à 447 000 acquéreurs, soit 8 % du total des allocataires en 2016, pour un montant moyen de 155 euros mensuels. L'APL-accession constitue donc un exemple d'utilisation maîtrisée des dépenses publiques et économiques, puisque le montant moyen est inférieur aux APL locatives- environ 260 euros par mois -, ce qu'a par ailleurs confirmé la Cour des comptes dans son rapport public d'octobre 2016, en reconnaissant la pertinence de ce dispositif qui permet de diminuer de 1,7 à 2 points le taux d'effort des ménages accédant Enfin, il y a, selon moi, une absence de vue du Gouvernement, qui souhaite supprimer ce dispositif, alors même qu'il veut aussi s'attaquer aux « passoires thermiques », ces logements mal isolés énergivores. effet, les prêts d'accession sociale et les prêts conventionnés peuvent aussi financer certains travaux d'agrandissement ou d'amélioration du logement, d'adaptation aux besoins d'une personne en situation de handicap ou d'économies d'énergie. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble de mes collègues à voter en faveur de l'amendement de suppression de l'article 52. La parole Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences de l'article 52 de la loi de finances pour 2018 sur les territoires dits détendus, et plus particulièrement sur les territoires ruraux comme celui dont je suis issu, la Nièvre. Dans ces territoires détendus, la réduction de loyer de solidarité, la RLS, pour les locataires du parc social, corrélée à une baisse du montant de l'APL calibrée de telle façon que la baisse de l'aide soit toujours inférieure à la baisse de loyer, aura un effet antipéréquateur. Dans nos territoires dits détendus, pour des raisons tant sociales, les locataires ayant de très faibles revenus, qu'économiques- le marché tire vers le bas les loyers au regard de la concurrence entre le secteur public et le secteur privé -, l'APL n'a pas pour effet, à la différence des territoires tendus comme Paris ou la région parisienne, de tirer les loyers vers le haut. Bien au contraire, sur nos territoires, la mise en oeuvre du prélèvement sur les bailleurs sociaux plus grande difficulté que ceux qui sont situés sur le reste du territoire. À titre d'exemple, compte tenu de leurs politiques de loyers actuelles et d'un dispositif RLS reposant sur un montant

De plus, en affaiblissant les capacités d'investissement des organismes d'HLM, cet article met en grande difficulté le secteur économique local du bâtiment. En effet, les pertes en exploitation ne permettront plus aux bailleurs sociaux de dégager un autofinancement indispensable à la mise en oeuvre de leurs opérations d'investissement. Selon les données de l'Union sociale pour l'habitat pour la région Bourgogne-Franche-Comté, avec cette mesure, ce seront 4 200 logements qui ne seront pas réhabilités et plus de 420 millions d'euros de travaux qui ne seront pas engagés avec, pour conséquence, 6 000 emplois détruits par an. En définitive, si le projet de loi de finances 2018 n'intègre pas de modalités spécifiques aux territoires ruraux en reconnaissant leurs particularités, les organismes locaux présents sur ces territoires dits détendus seront voués à disparaître au profit d'une concentration et de regroupements dont il n'est pas démontré qu'ils auront une connaissance aussi fine des besoins locaux et qu'ils sauront participer au mieux à la réhabilitation des centres-bourgs et des centres-villes, dont l'urgence est patente. Monsieur le ministre, est-ce la mort de nos organismes locaux sans discernement sur leur efficacité et la pertinence de leur action qui est ici visée ? La parole

140 euros n'iront pas à l'entretien de l'immeuble, encore moins à l'entretien des espaces collectifs et aux services rendus aux locataires. Et voici que l'article 52 met en question les aides personnelles au logement, qui intéressent la majorité des locataires du parc social, puisque 60 % de ceux-ci disposent de ressources inférieures à 60 % des plafonds de ressources. Dans les faits, les populations les plus modestes, que leur revenu situe dans les 30 % les moins riches de la population, constituent une proportion deux fois plus importante des familles logées en HLM. Autant dire que la mise en place du prélèvement forfaitaire unique ne représente quasiment rien pour elles, pas plus que la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, et la réforme de la taxe d'habitation peut en laisser certains de bois Par contre, l'article 52 les concerne tout de suite ! Car voilà un article qui, au nom de l'équilibre des comptes publics et du juste partage des efforts, vient demander à des familles très majoritairement modestes, probablement d'ailleurs dispensées du paiement de l'impôt sur le revenu et de tout ou partie de leur taxe d'habitation, d'apporter rien de moins que 720 euros par an au titre de la baisse de l'allocation, soit 1,7 milliard d'euros par an pour le secteur ... Le tout en échange d'une baisse quasi artificielle des loyers, dont la conséquence principale sera d'assécher les fonds propres des organismes bailleurs. Résumons ! Nous avons, d'un côté, une opération de baisse des allocations, une baisse des loyers dans le secteur social conventionné, qui mettra en voisinage des familles allocataires à taux d'effort constant et des familles non allocataires à taux d'effort allégé, et, de l'autre, des organismes bailleurs qui n'auront plus les moyens d'entretenir correctement leur patrimoine ni, surtout, d'autofinancer sur leurs fonds propres quelque opération de réhabilitation de logements ou de construction neuve que ce soit. que ce soit. Quoi qu'il arrive, le Gouvernement met le secteur du logement social dans la plus grande difficulté quant à sa participation réelle au nouveau programme national de renouvellement urbain. L'article 52 pose le problème récurrent de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, puisque la baisse des loyers accompagnant celle des allocations profitera autant aux allocataires qu'aux autres. De plus, il crée des conditions de financement des organismes de logement social social extrêmement périlleuses pour ces organismes eux-mêmes, mais aussi pour le secteur d'activité du bâtiment- on a parlé de fonds de roulement ; parlons clair : le logement social, c'est des « fonds de roulement » pour le BTP

par le niveau de la baisse des loyers. Dès lors, comment trouverons-nous les financements nécessaires au lancement de nouveaux programmes ? Comment poursuivrons-nous l'amélioration de l'existant ? Comment répondrons-nous aux milliers de foyers inscrits sur nos listes d'attente ? Ce ne sont pas des mots ni des propos de tribune prétendument alarmistes ; ce sont des faits, uniquement des faits

hauteur de 400 millions d'euros, des recettes que nous n'avons pas voulu avoir. En revanche, on a doublé la valorisation des stock-options, et on a doublé l'amélioration des aides fiscales pour les impatriés des multinationales.

le bâtiment. Non, les APL ne sont pas inflationnistes ! Elles l'ont été dans les années 1995 à 2000 ; mais elles ne le sont plus aujourd'hui.

de logement, mais les aides au logement ne représentent que 0,9 % du PIB depuis 1996. Ce qui a dérapé dans les dépenses, ce n'est pas l'APL Ce sont les aides fiscales, toute une autre série d'aides qui méritent d'être évaluées. Oui, pas d'immobilisme ! Oui, il faut repenser une autre politique du logement ! Sans doute y a-t-il de la déperdition ici ou là

La parole est à Mme Viviane Artigalas,

l'APL-accession, 450 000 ménages modestes ont pu acquérir leur logement, pour une enveloppe de 800 millions d'euros par an. L'étude toute récente du Crédit foncier rappelle que ces ménages ont acheté pour 33 % d'entre eux et 77 % dans l'ancien, et ces acquisitions ont concerné majoritairement les zones détendues. L'APL-accession permet donc l'accès à la propriété de ménages aux revenus modestes, particulièrement dans les centres-bourgs et parfois dans des zones où il n'y a pas d'offre locative adaptée pour ces familles. Dans de nombreux cas, le projet d'acquisition n'aurait pu être possible sans le soutien de l'APL-accession, qui intervient comme un réel déclencheur, même s'il est moindre que celui du prêt à taux zéro. Par ailleurs, l'APL-accession est souvent nécessaire pour conforter un prêt aidé. Pour les ménages du premier quartile bénéficiant d'un prêt à taux zéro, elle permet de réduire d'un quart les mensualités de remboursement. En termes d'économies budgétaires, l'intérêt de la suppression de cette aide est nul sans APL-accession, les ménages se maintiennent dans le parc locatif et continuent donc de bénéficier de l'APL locative. La suppression voulue par le Gouvernement est bien contre-productive, car elle aura pour effet de bloquer la mobilité des ménages les plus modestes, sans créer, pour autant, d'économies importantes pour l'État. Elle n'est pas non plus cohérente avec les objectifs énoncés par le Président de la République, à savoir rendre 40 000 locataires de logements sociaux propriétaires de leur habitation. Comment voulez-vous rendre 40 000 ménages propriétaires sans aides, alors que, pour la plupart d'entre eux, ils n'en ont pas les moyens ? Enfin, en soutenant ces ménages, on soutient l'activité du bâtiment, qui se serait sans doute effondrée dans certains territoires sans les aides publiques. Vouloir supprimer l'APL-accession est donc une grave erreur, car cela aura des répercussions à long terme, non seulement sur les familles, mais aussi sur l'activité économique de nos départements. Et je doute que le Gouvernement les ait bien mesurées avant de prendre une telle décision

le mouvement HLM est profondément déstabilisé par la soudaineté et la brutalité des mesures non concertées de ponction directe sur les recettes des organismes annoncées par l'État. La mobilisation de l'ensemble des acteurs du logement est forte pour protester contre les conséquences désastreuses de cette politique sur le développement de l'habitat social, les politiques locales de l'habitat et l'emploi local. Les pertes de recettes pour les bailleurs sociaux dans la région des Hauts-de-France sont estimées à 233 millions d'euros par an, ce qui les conduirait inéluctablement à stopper leurs investissements 1,4 milliard d'euros de travaux en moins, 13 500 logements rénovés en moins et 19 200 emplois directs et indirects menacés dans la région des Hauts-de-France. Sera particulièrement touché dans mon département du Pas-de-Calais le patrimoine minier : des logements mis à disposition des mineurs et de leurs familles au temps de l'exploitation charbonnière et repris aujourd'hui par un bailleur qui n'a de cesse de les rénover et de les rendre plus confortables pour les proposer à nos populations. Il en est de même pour le premier bailleur social de mon département, Pas-de-Calais habitat, dont la politique de rénovation et de construction de logements sera fortement ralentie, mettant en péril la qualité de l'offre locative et l'emploi induit dont a cruellement besoin notre territoire. Ce n'est pas au logement social et à l'APL, coeur de la solidarité nationale, de contribuer, en première ligne, à cet effort. Vous attaquez, une fois de plus, les classes moyennes et populaires, alors même que vous supprimez l'impôt sur la fortune. Des compensations sont, certes, en discussion, mais il est à craindre que ces compromis ne soient ni satisfaisants ni efficaces et qu'ils ne permettent pas d'atteindre les objectifs du Gouvernement : choc de l'offre, moins de sans-abri, moins de frais de gestion. C'est pourquoi nous souhaitons la suppression pure et simple de l'article 52 du projet de loi de finances pour 2018. d'État, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'économie générale de l'article 52 : nous sommes presque tous d'accord ici pour dire qu'il

C'est la raison pour laquelle de nombreux collègues ont déposé des amendements, notamment en commission des finances, pour tenter de manière transpartisane de le faire évoluer. C'est en ce sens que le groupe socialiste et républicain a déposé un certain nombre d'amendements, qui ont eu le bonheur d'être

Cela signifie que les populations les plus défavorisées- je ne mentionne pas les indicateurs socio-économiques -vont participer à l'effort de ceux qui sont déjà un peu mieux lotis.

Je m'étonne de l'obsession du Gouvernement sur le coût du logement pour l'État : il ne voit cette politique que comme une charge, en niant que la construction de logements est

emplois menacés. Sans compter la perte de recettes fiscales, d'environ 600 millions d'euros. Je puis comprendre la volonté de réforme du Gouvernement ; à titre personnel, je n'y suis pas hostile. Mais, enfin,

angulaire du système HLM. C'est pourquoi le Sénat a cherché une solution de compromis, qui permette de réaliser l'économie budgétaire demandée par le Gouvernement sans toucher au loyer et, en conséquence, sans déstabiliser le secteur HLM. J'espère, monsieur le ministre, que le Gouvernement entendra cette démarche.

tout de même que les taux de loyers appliqués dans le logement social sont réglementés et plafonnés, que le parc public accueille un ménage sur deux en dessous du seuil de pauvreté, que près de 150 000 logements sociaux ont été programmés en 2017 et que les organismes réinvestissent leurs marges dans ces opérations.

Plus de 50 % des organismes HLM pourraient se retrouver rapidement dans une grave difficulté financière ! Quant aux collectivités territoriales,

on abandonne la progressivité, on prend les 800 millions d'euros sur 2018 et 2019 et on se revoit après l'engagement de la réforme structurelle, je crains que nous n'en sortions pas ! À ce moment-là, toutes les heures que nous avons passées pour essayer

J'ai souhaité que l'on puisse introduire de la TVA dans le système, parce que j'étais convaincu depuis le début que c'était une bonne initiative- comme on pouvait aussi réfléchir sur la question des charges et un certain nombre d'autres sujets. Nous avons donc

rectifié. L'article 52 réformerait de manière drastique les aides au logement et les loyers dans le parc social. En effet, plus le bailleur social logerait de personnes modestes, plus il serait taxé ; plus la famille serait nombreuse, plus la taxe serait élevée. Cette mesure est contraire à l'esprit du logement social.

d'une réforme globale des aides au logement, le Gouvernement fait le choix d'un changement à la marge qui risque de pénaliser durement les bailleurs. La baisse annoncée des APL sera répercutée directement sur les bailleurs, qui devront baisser d'autant leurs loyers. Ces mesures vont engendrer un affaiblissement évident des bailleurs sociaux ; elles auront probablement un impact sur le nouveau programme national de renouvellement urbain et mettront en péril les engagements financiers des bailleurs pour prendre en charge la réhabilitation et la construction de nouveaux logements. À cela s'ajoute la suppression des APL-accession, qui réduira nécessairement la capacité des ménages à accéder à la propriété. Nous faisons également observer que la décision d'appliquer le surloyer de solidarité dès le premier euro de dépassement du plafond pénalisera, une fois de plus, les bailleurs. Plutôt que de remplir le rôle compensatoire, il aura l'effet inverse. En cas de départ d'un locataire pour cause de supplément de loyer de solidarité, il sera remplacé par un locataire bénéficiaire des APL dont la baisse sera compensée par bailleur. Pour toutes ces raisons, j'invite le Sénat à supprimer l'article.

Ainsi, sous couvert de réduire la part de l'État dans le financement des APL, l'article 52 en transfère la charge sur les bailleurs sociaux. Or ceux-ci sont particulièrement sollicités, par ailleurs, pour le financement de la politique de la ville- à hauteur de 2 milliards

Enfin, le Sénat a adopté une augmentation de la TVA sur la construction de logements sociaux qui devrait rapporter à l'État plus de 600 millions d'euros. Ces mesures vont directement pénaliser la construction et la réhabilitation de logements sociaux, d'une manière ou d'une autre. ce sont les bailleurs, donc les locataires, qui financeront pour partie les aides au logement, ce qui ne correspond pas à notre vision de la solidarité nationale. À l'inverse, et alors que les loyers du secteur privé s'envolent, vous ne faites rien pour limiter le poids public des APL. Deux poids, deux

d'un secteur qui le réinvestit pourtant intégralement dans la production et la réhabilitation de logements locatifs sociaux. S'agissant des contreparties que vous proposez, monsieur le ministre, elles sont inquiétantes. Vous proposez en effet aux offices HLM d'emprunter toujours plus. Vous leur proposez également de vendre le patrimoine, au moment même où la file des demandeurs

avec un loyer moyen de 390 euros, contre 570 euros dans le parc privé, les organismes HLM répondent à une demande sociale forte. Outre la brutalité de la mesure proposée, est difficile d'accepter que l'effort de réduction budgétaire continue à toucher les plus pauvres. C'est totalement contradictoire avec la volonté affichée du Gouvernement de demander aux offices HLM de loger encore plus de personnes démunies, comme en témoigne votre projet Logement d'abord. le résultat d'exploitation des organismes HLM, 2,2 milliards d'euros annuels, est intégralement réinvesti dans la production de logements et la rénovation du parc, avec des effets démultiplicateurs en termes d'activité, d'emplois directs et indirects et de TVA à hauteur de 800 millions d'euros ? La baisse des APL revient à prélever sur les organismes HLM 1,7 milliard d'euros en 2018, amputant ainsi leur capacité d'investissement de 75 %. Plus d'une centaine d'organismes HLM seront mis en péril, alors que plus d'une centaine d'autres connaîtront les plus grandes difficultés. Ces organismes sont présidés par des élus locaux, notamment des maires, ce que l'on ne saurait oublier.

coûteuses à mettre en oeuvre et, bien sûr, évolutives à la hausse par l'effet de paupérisation des locataires des quartiers dont on connaît la réalité au sein du parc public. Plus le parc se paupérisera, plus les offices HLM seront taxés ! C'est pourquoi le groupe socialiste et républicain propose la suppression de l'article 52.

en l'état. Cependant, j'attends avec impatience la réponse du ministre sur la situation des outre-mer. En tout cas, le sort qui leur est infligé n'est pas acceptable

d'accession très sociale et d'amélioration lourde de l'habitat, ainsi que de 300 ventes de logements locatifs à leurs locataires par an. Cette mesure affecterait fortement le BTP, secteur déjà très en crise, et donc les emplois, avec une baisse de 45 millions d'euros d'investissement par an. Elle aurait également des effets négatifs considérables sur toutes les thématiques d'aménagement urbain durable, sur les objectifs d'acquisition urbaine de la nouvelle politique de la ville, sur les projets d'action sociale de mixité et de diversité de l'habitat, sur la lutte contre l'habitat indigne et insalubre, et sur le maintien de la solidarité des familles et la stabilité sociale à la Réunion. Aussi irai-je dans le même sens que mes collègues. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

Le scrutin est ouvert.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

j'ai le plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de la commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse et de l'enfance de l'Assemblée nationale vietnamienne, conduite par son président, M. Phan Thanh Binh. La délégation est accompagnée de notre collègue Catherine Deroche, présidente du groupe d'amitié France-Vietnam. La France et le Vietnam s'apprêtent à célébrer en 2018 un double anniversaire : quarante-cinq ans de relations diplomatiques bilatérales et cinq ans de partenariat stratégique. La France a été l'un des premiers pays occidentaux à soutenir la politique de rénovation du Vietnam et à accompagner le développement et l'ouverture de ce pays. La délégation échangera demain avec plusieurs sénateurs de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication présidée par Mme Catherine Mme Catherine Morin-Desailly, pour évoquer les coopérations universitaires et scientifiques entre nos deux pays et la préparation des Jeux de l'Asie du Sud-Est que le Vietnam accueillera en 2021, alors que Paris accueillera les jeux Olympiques en 2024. En votre nom, mes chers collègues, je leur souhaite de fructueux travaux, espérant que ce séjour permette de renforcer nos relations avec le Vietnam, et de donner un nouvel élan à la francophonie, au sein de la jeunesse en particulier.

Quel est l'avis du Gouvernement ? votre amendement. Le rapporteur Philippe Dallier a parlé de constance. Moi, je salue la fidélité à vos convictions.

du taux de TVA sur les investissements réalisés par les bailleurs sociaux sur les constructions et les rénovations de logements sociaux. Le rendement de cette

par les bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social, et cela à hauteur de 850 millions d'euros. Nous porterions ainsi le taux de la cotisation dite « cotisation principale à 7 %. Par ailleurs, l'article 52 auquel vous avez fait référence, monsieur le ministre, supprime le dispositif d'APL-accession, au motif que ce dispositif serait peu pertinent et peu attractif. Or je me permets de vous rappeler que la Cour des comptes, dans son rapport de novembre 2016 sur les aides de l'État accordées pour l'accession à la propriété, a souligné que c'est parce que les conditions d'accès à l'APL-accession sont devenues particulièrement restrictives qu'elles excluent, de fait, un nombre important d'accédants, alors même que leur effet solvabilisateur est utile aux ménages. Je rappelle également que les économies attendues de la suppression du dispositif APL-accession sont particulièrement faibles : 50 millions d'euros. En outre, cette disposition n'intègre pas du tout les coûts supplémentaires liés au fait que certains ménages qui pourraient ne pas accéder à la propriété continueraient de fait à recevoir les aides personnelles au logement. Le Sénat, vous le savez, s'est déjà opposé à une telle suppression de l'APL-accession lors de l'examen

Vous pourriez vous demander pourquoi nous ne sommes pas parvenus à un amendement commun. Tout d'abord, les amendements ont été rédigés à une semaine d'intervalle. Celui de la commission des affaires économiques a été rédigé pour le mercredi suivant l'examen de la première partie

que j'ai présenté cet amendement en commission des finances. Pourquoi ai-je la faiblesse de croire que celui-ci est meilleur ? C'est parce que je suis persuadé qu'il est sur le chemin du compromis qui finira par être trouvé

certes pas le seul -de soutien aux parcours résidentiels. L'APL-accession représente une part très réduite des APL : 5 % des 18 milliards d'euros, soit 800 millions d'euros par an. Elle concerne environ 450 000 ménages, pour un montant moyen de 155 euros par mois.

Dans un rapport rendu public en novembre 2016, la Cour des comptes reconnaissait la pertinence de ce dispositif, qui permet de diminuer de 1,7 à 2 points le taux d'effort des ménages. Cette suppression nuira donc grandement à la capacité des ménages aux revenus modestes et moyens d'accéder à la propriété, tout en aggravant, à court terme, le déficit public. En effet, si l'effet déclencheur de l'APL-accession est moindre que celui du PTZ, il est réel, et aura d'autant plus le présent projet de loi de finances tend à réduire, à plus ou moins long terme, les périmètres géographiques d'application du PTZ. Ainsi, 65 % des bénéficiaires de l'APL-accession résidant en zone 3, l'équivalent de la zone C pour le parc privé, soit la zone où le PTZ sera supprimé. année, 23 000 ménages pourraient donc être privés, non seulement de la solution de l'accession sociale, mais aussi du prêt à taux zéro dans ces mêmes zones C. Ce sont, au final, autant d'opérations qui ne seront probablement pas réalisées, ce qui représentera une perte de recettes pour l'État nettement supérieure

réduira ainsi la mutation dans le parc social et la mobilité, que le Gouvernement appelle pourtant de ses voeux. Le présent amendement tend donc à la supprimer.

En réduisant leur taux d'endettement, ces aides soumises à des conditions de revenus permettent à des ménages modestes de devenir propriétaires de leur résidence principale, alors qu'ils ne pourraient pas souscrire un prêt immobilier autrement. aides ne sont pas inefficaces. La Cour des comptes leur en a en effet reconnu, dans un rapport publié en novembre 2016, un réel effet redistributif, bien qu'elle recommande une nécessaire rationalisation des aides de l'État en matière d'accession à la propriété. La suppression de ces aides pour une économie annuelle de 50 millions d'euros est, notamment, un mauvais signal donné à la jeunesse, qui peine à accéder à la propriété. Au lieu d'être définitivement écarté, ce dispositif mériterait d'être renforcé. L'amendement

à mettre en place une réduction de loyer de solidarité, dite RLS, pour les locataires du parc social, établie en fonction de la composition du ménage et s'appliquant pour les ménages en deçà d'un certain plafond de ressources. La RLS compenserait une diminution de l'aide personnalisée au logement pour les bénéficiaires locataires du parc social, diminution équivalente à une fraction comprise entre 90 % et 98 % de cette Cette réduction de loyer de solidarité pénaliserait lourdement les organismes majoritairement détendeurs d'un parc à bas loyer construit avant la création des allocations personnalisées au logement de 1977. En effet, ce parc requiert des investissements très lourds en matière de réhabilitation, en raison de sa vétusté. Aussi, il faut préserver les recettes des organismes sur ce patrimoine, afin que ceux-ci puissent procéder aux importantes opérations de réhabilitation qui Par ailleurs, il n'est pas pertinent de soumettre l'offre nouvelle à bas loyer à cette baisse de l'APL et à cette RLS. L'offre en prêts locatifs aidés d'intégration dans le neuf, dont les loyers sont calculés en optimisant les loyers plafonds APL, doit être exemptée de ces mesures, car elle est nécessaire à la mise en oeuvre de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté pour déspécialiser les quartiers fragiles. Dans un parc à bas loyer, dans l'ancien comme dans le neuf, l'exonération de la baisse des APL et, donc, de la RLS permettra de ne pas fragiliser les offices qui accueillent le plus grand nombre de ménages modestes. organismes pourront ainsi mettre en oeuvre une politique de rééquilibrage des locataires, qui les incitera à produire davantage de logements destinés à l'accueil des ménages modestes. La stabilité des recettes provenant des loyers est à la base du modèle de gestion du logement social, et cela afin d'amortir l'ensemble des emprunts souscrits.

du dispositif de péréquation, donc de mutualisation financière, les organismes de logements sociaux des départements et collectivités d'outre-mer.

touche autant à la mixité sociale qu'à la politique des loyers et à la réforme du secteur HLM. Mais je veillerai, et je le dis très clairement devant le Sénat, à ce que la question de l'APL-accession soit à nouveau

Si le Gouvernement, et je le dis aussi très clairement, partage l'objectif de protéger les bailleurs les plus sociaux, en leur donnant les moyens suffisants, deux mesures proposées soins vont déjà dans ce sens. La première est l'exclusion de l'ensemble des logements-foyers et des organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion du champ de l'article 52-

Il faut conclure, mon cher collègue.

parlementaire où des oppositions, de natures pourtant très différentes, tentent de trouver une solution face à un gouvernement qui s'est enferré, cet été, dans des propositions expéditives.

Au détour d'une mesure budgétaire, certes nécessaire, nous avions le sentiment qu'il existait des voies de passage différentes, associant l'ensemble des acteurs qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice,

le groupe socialiste s'oppose à la baisse des aides au logement dans le parc social. Il regrette que le Gouvernement continue sa politique d'économies sur le logement social. En baissant drastiquement le montant des aides au logement du parc social, le Gouvernement affaiblit les organismes HLM.

Le groupe socialiste, comme il l'a fait en commission des affaires économiques, votera l'amendement n° II-285 de Mme Estrosi Sassone déposé au nom de la commission. Il s'agit

nous considérons malheureusement que c'est la seule alternative envisageable à la décision du Gouvernement de baisser de 1,5 milliard d'euros les APL dans le parc public et de mettre en place, en compensation, une réduction du loyer de solidarité appliqué par les bailleurs. Nous le répétons, pour nous, la baisse des APL et la réduction du loyer de solidarité ne sont pas des solutions de compromis. L'amendement n° II-285 est le seul amendement qui correspond au compromis

a déjà fait beaucoup dans la négociation avec les bailleurs, nul ne l'a rappelé ici. Il a introduit une progressivité sur trois ans pour atteindre l'objectif de 1,5 milliard d'euros. C'est une première concession. des compensations de l'ordre de 700 millions d'euros, les 800 millions d'euros restants doivent être trouvés par des économies de gestion et de restructuration sur trois ans. Une stabilisation du taux du Livret A correspondant à une baisse des charges financières de l'ordre de 700 millions d'euros par an, une enveloppe additionnelle de 2 milliards d'euros de prêts à des taux de bilan bonifiés, un allongement de la maturité des prêts aux bailleurs sociaux qui devrait produire un gain de trésorerie de 250 millions d'euros

Vous représentez le mouvement gaulliste : heureusement qu'à une époque le Sénat de la République s'est opposé au Gouvernement ! Parce que nous ne commettons pas, nous, de forfaiture et respectons la Constitution, ce qui n'était pas forcément le cas ; le président Monnerville avait bien raison à l'époque. D'ailleurs, ensemble, cher président Retailleau,

est d'accord avec les propositions du Gouvernement. C'est une réalité, l'avenir proche le démontrera.

Le scrutin est ouvert.

: extraire de la cotisation principale, dont le produit est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social, le supplément de loyer de solidarité

Quel est l'avis de la commission ?

je suis effectivement défavorable à cet amendement, qui exclut de l'assiette de la cotisation principale versée par les bailleurs

cet amendement majore les recettes affectées au Fonds national d'aide au logement de 150 millions d'euros et augmente les dépenses du Fonds de 850 millions d'euros, dont 400 millions d'euros liés à une moindre économie due à la réduction de loyer de solidarité et 50 millions d'euros au maintien de l'APL-accession. Quel est l'avis de la commission ?

Les maires des villes fortement engagées dans la politique de la ville se sont réunis lors d'états généraux en octobre dernier. Ils ont dressé un constat sur les urgences qui menacent aujourd'hui un certain nombre de quartiers prioritaires. Ils ont aussi proposé un projet commun avec des politiques correctives et des moyens financiers dédiés. L'appel de Grigny » lancé au Président de la République a donc été l'occasion d'alerter sur la situation critique des quartiers et de leurs habitants, mais aussi de proposer des mesures d'urgence. La création d'une plateforme nationale des initiatives issues des quartiers, d'un réseau accélérateur de ces initiatives et d'un fonds de développement de 100 millions d'euros figure parmi les dix mesures d'urgence à mettre en oeuvre. Le Président de la République veut faire des quartiers de la politique de la ville de « grands territoires gagnants Il s'est engagé dans son discours de Tourcoing, le 16 novembre dernier, à encourager l'ensemble des acteurs et les associations qui jouent un rôle fondamental dans les quartiers : il a annoncé la mise en place d'une plateforme mettant en ligne les bonnes initiatives et permettant de les financer pour les démultiplier dans démultiplier dans tous les territoires où elles sont pertinentes. Les associations locales font souvent mieux que les pouvoirs publics et c'est le rôle de l'État de contribuer à leur financement. Le Président de la République a parlé de « plan de bataille ». Allons-y : les quartiers sont prêts et n'attendent que cela 100 millions d'euros pour lancer cette bataille, pour redonner confiance et espoir aux 5 millions d'habitants qui vivent dans les quartiers les plus en difficulté, 100 millions d'euros pour asseoir la crédibilité du discours du Président de la République et contribuer à la grande mobilisation nationale annoncée. suggérons au Gouvernement la création sans délai d'une plateforme nationale intitulée Agence des solutions locales. L'objectif est d'accorder le soutien des acteurs économiques, des collectivités et des services de l'État aux initiatives locales participant à l'amélioration de la vie des habitants. Notre amendement prévoit de doter cette agence, dès 2018, de 100 millions d'euros de crédits dédiés au portage des initiatives issues des quartiers. Au regard des engagements pris par le Président de la République de soutenir les projets innovants à forte utilité sociale et compte tenu de l'urgence à intervenir, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission soient majorés en conséquence par le Gouvernement, sans faire supporter cet effort à un autre programme de la mission.

la politique technique et la qualité de construction, mais aussi 20 millions d'euros sur l'urbanisme et l'aménagement, au programme 135, ce qui réduirait très fortement les moyens mobilisés par l'État

Mais, attention : le projet de renouvellement urbain s'étale dans la durée, alors qu'il nous faut répondre sans délai aux préoccupations des habitants des quartiers de la politique de la ville, notamment en matière d'emploi, de sécurité, d'offre éducative et d'équipements ... Or le budget pour 2018 prévoit pour le financement de l'ANRU 15 millions d'euros en crédits de paiement et 15 millions d'euros en Cela signifie qu'il ne se passera rien en 2018 et en 2019 ! Deux années perdues, monsieur le ministre ! Les habitants des quartiers ne vont pas le comprendre. Même si nous sommes encore en phase de préfiguration pour le NPNRU,

Au regard des engagements pris par le Président de la République envers les quartiers et leurs habitants dans le cadre de la grande mobilisation annoncée dans son discours de Tourcoing, il apparaît nécessaire que le Gouvernement majore les crédits de l'ANRU sans faire supporter cet effort à un programme de la mission.

Cette aide, mise en place dès 2015, répondait à une demande forte de l'ensemble des élus locaux, notamment de l'Association des maires de France. Le Gouvernement vient de supprimer cette aide. Soutenir les communes qui font les efforts nécessaires pour améliorer l'accès au logement de nos concitoyens nous paraît pourtant essentiel. Cet amendement prévoit donc de rétablir pour 2018 les crédits de l'aide aux maires bâtisseurs à hauteur

et fixer un objectif de 10 000 logements accompagnés par an sur 3 ans, en commençant par 4 000 cette année, pour une dépense de 14 millions d'euros. Vous en conviendrez, monsieur le ministre, ce n'est pas une ruine pour l'État

sujet. Quel est l'avis de la commission ?

Les moyens dégagés en 2018 vont permettre de répondre à l'ambition du plan Logement d'abord. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il est hors de question d'utiliser les crédits dédiés à l'hébergement d'urgence

de projets créateurs d'emplois et d'activités durables dans les zones prioritaires. Le présent amendement vise à transférer une partie des crédits de l'action n° 07, Urbanisme et aménagement, du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », à hauteur de 5 millions d'euros, vers l'action n° 01, Attractivité économique et compétitivité des territoires, du programme 112 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ». Cette augmentation des autorisations d'engagements allouées en 2018 à la prime d'aménagement du territoire permettra de revenir au même budget alloué à la prime d'aménagement du territoire qu'en 2017, soit 20 millions d'euros. La parole

Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits, modifiés. Mes chers

une pénurie de services publics. Cet amendement vise uniquement à commander au Gouvernement un rapport d'information sur l'opportunité de créer un indicateur d'évaluation de la présence des services publics et parapublics dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans ces zones rurales, ni plus ni moins.

ont élaboré des outils indicateurs, des cartes des données territoriales, qui permettent d'estimer la disponibilité des services et le temps d'accès de la population. Je veux bien qu'on commande un nouveau rapport, mais reste à savoir s'il sera déposé. Le Parlement